est à M. Guillaume Arnell. Lors du scrutin n° 127 sur l'amendement n° 712 rectifié, MM. Joël Labbé et Roland Dantec ont été enregistrés comme ayant voté contre, alors qu'ils souhaitaient voter pour. Par ailleurs, lors du scrutin n° 129 portant sur les amendements identiques n 1 rectifié, 542 rectifié et 762 rectifié, MM. Joël Labbé et Jean-Marc Gabouty ont été enregistrés comme s'étant abstenus, alors qu'ils souhaitaient voter pour.

politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

Le présent amendement prévoit que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, tels que les 1 300 médecins généralistes de SOS Médecins France, puissent avoir toute leur place et être agréés maîtres de stage pour accueillir au sein de leur structure des étudiants, afin qu'ils puissent compléter leur formation

rectifié est effectivement satisfait, puisque les textes encadrant la formation de troisième cycle des études de médecine prévoient les conditions d'octroi par l'ARS, sur proposition des facultés de médecine, des agréments permettant d'accueillir les internes en stage. Ils sont délivrés sur la base du projet pédagogique qui peut être proposé par le médecin généraliste aux internes qui réaliseraient un stage sous son encadrement. La proposition d'accueil d'étudiants au sein des associations de PDSA est tout à fait possible en l'état actuel du droit. C'est donc, dans les faits, la présentation de projets pédagogiques par ces maîtres de stage et les demandes d'agrément déposées auprès des facultés de médecine qui permettront à l'ensemble de ces stages de se matérialiser. Le Gouvernement demande donc le retrait de

afin que les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur continuent de fixer le nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision territoriale. En effet, certaines spécialités, notamment la gynécologie médicale- mais il en existe certainement d'autres -souffrent d'un manque d'effectifs. Il existe ainsi un risque, pressenti par les professionnels, d'extinction de la discipline.

régionaux. La responsabilité des universités à l'égard des départements qui les entourent est insuffisamment énoncée. L'université ne peut plus continuer de former des médecins sans se préoccuper de leur exercice dans les départements. L'amendement

Je m'interroge sur la notion de représentants de la profession dans les territoires et celle de représentants de la profession dans les départements. Elles me paraissent beaucoup trop imprécises pour figurer dans la loi. De qui s'agit-il exactement ? En tout état de cause, j'espère que les professionnels seront en effet consultés pour la détermination des postes d'internat, sans qu'il soit

les professionnels du secteur, est prévue. Par conséquent, les acteurs du système de santé et des formations médicales sont représentés dans cet observatoire régional. Je l'ai dit hier, nous pensons qu'il faut renforcer le pilotage de ces structures, qui évaluent la démographie médicale et les besoins en professionnels de santé.

et 50 % des Guyanais diplômés du supérieur partent y chercher un emploi. Il y a là un sérieux problème pour le développement économique de ces territoires, qui vivent une véritable fuite des cerveaux, alors même que le taux de diplômés du supérieur y est encore inférieur à celui de l'Hexagone. La situation sociodémographique des outre-mer conduit à un paradoxe spécifique alors que les besoins en offre de soins y sont en moyenne plus élevés, l'accès aux soins y est rendu plus difficile. Cela tient évidemment au départ de nombreux jeunes médecins, mais aussi au vieillissement croissant de la population.

rappelé devant l'Assemblée nationale qu'il n'existait pas encore de cursus d'études de médecine complet dans ces territoires. Les étudiants sont donc obligés de partir effectuer leur deuxième cycle ailleurs, ce qui réduit de fait leurs chances d'exercer la spécialité de leur choix dans leur région d'origine.

L'alinéa 10 prévoit en effet que l'affectation des étudiants sur les postes d'internat tient notamment compte du parcours de formation antérieur et du projet professionnel des étudiants.

Notre rôle de parlementaires est de nous attaquer à ce problème et de permettre à chacun de pouvoir se soigner quel que soit son lieu de résidence, et ce dans les meilleures conditions possible. Or force est de constater que le présent projet de loi ne répond

nous proposons une piste intéressante pour inciter les étudiants en médecine à effectuer des stages en zones sous-denses et à venir ainsi renforcer l'offre de soins dans les territoires les moins bien dotés. moins bien dotés. L'accès au troisième cycle de médecine est conditionné par l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis des connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Les étudiants sont ensuite répartis sur des postes ouverts par spécialité et par subdivision territoriale. Leurs choix sont satisfaits ou non en fonction de leur classement, qui prend en compte leurs résultats aux épreuves, leur parcours de formation, leur projet professionnel et, le cas échéant, leur situation de handicap.

devrait être prépondérant.

les résultats à des épreuves spécifiques de compétences et de connaissances, auxquelles les étudiants devront avoir obtenu une note minimale, le parcours de formation des étudiants, leur projet professionnel, ainsi que, le cas échéant, leur situation de handicap. Animé par la même inquiétude que les auteurs amendements, j'ai interrogé la DGOS sur la hiérarchisation de ces différents critères. Elle m'a indiqué que les résultats aux épreuves de compétences et de connaissances continueront de tenir une place prépondérante pour l'orientation des étudiants en troisième cycle ; je l'ai d'ailleurs écrit dans mon rapport. Mme la ministre pourra sans doute nous le confirmer. Il me semble donc inutile d'intégrer ces précisions dans la loi, d'autant que la rédaction des amendements pose plusieurs problèmes-

Quel est l'avis du Gouvernement ? La rénovation profonde des modalités d'accès aux études, manifestée notamment par la suppression des épreuves classantes nationales, ne signifie évidemment pas l'abandon du principe d'égalité entre les candidats.

Ces textes détermineront également les procédures permettant d'organiser les épreuves de vérification des compétences en situation, qui, par nature, ne sauraient être écrites,

Les établissements publics de santé ont dû s'adapter à cette évolution. Or force est de constater une hétérogénéité entre les régions en matière de politique d'agrément, et donc de répartition. Les interventions des ARS ont été très variables, s'agissant notamment du recours aux dérogations au taux d'inadéquation. Il est aujourd'hui fondamental de revoir et de préciser les conditions de mise en oeuvre des réformes des études médicales et le rôle des différents acteurs, notamment des coordonnateurs et des sociétés savantes. Les établissements doivent également être mieux associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques, et à ce titre intégrer la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie,

davantage associés à la gouvernance et au suivi des réformes pédagogiques et, à ce titre, intègrent la Cnemmop.

Madame la ministre Frédérique Vidal, vous aviez répondu à notre collègue Pierre Dharréville que, « compte tenu du nombre, de l'importance et du caractère éminemment transversal des différentes réformes des études médicales en cours, [vous n'étiez pas] opposée à l'idée d'adapter le dispositif de gouvernance en vigueur pour assurer la représentation des parties prenantes directement concernées et l'articulation

La commission n'est pas favorable à cette précision, pour une raison de forme et une raison de fond. Pour ce qui est de la forme, je ne vois pas bien à quoi se réfère la notion de « gouvernance de la réforme

Notre travail a en effet permis de constater l'absence totale d'une telle formation aujourd'hui. Pourtant, de plus en plus de patients recherchent des soins à base de plantes, parfois sans en parler à leur médecin, n'est souvent pas formé pour répondre à cette demande et ne pense pas nécessairement à interroger le patient sur ses pratiques. Le médecin ne pourra donc pas prendre en compte les potentielles interactions médicamenteuses. De plus, de nombreuses plantes sont d'une et présentent un véritable intérêt pour la santé publique. Pour ne prendre qu'un exemple, certaines huiles essentielles diminuent la résistance des bactéries aux antibiotiques. Il est donc essentiel de développer la formation des médecins à l'usage des plantes

ou de prévoir que les étudiants de troisième cycle seront formés à ces thématiques ? Dans le premier cas, la question de la recevabilité financière de l'amendement se poserait.

Comment sommes-nous passés à côté d'une telle richesse ? Comment l'avons-nous ignorée, avec quelque mépris parfois pour des pratiques ancestrales qui avaient fait leurs preuves ? Comment avons-nous pu abandonner ces médications d'équilibre, aveuglés par le mirage du « tout chimique » Comment avons-nous pu supporter les effets secondaires des médicaments, dont les listes, longues comme le bras, sont éloquentes et font littéralement peur ? Bien sûr, la chimie est nécessaire, mais elle ne peut pas tout. Il faut le reconnaître, nous sommes allés trop loin en voulant remplacer ce qui était efficace contre les maux du quotidien. Les plantes sont notre chance ; nous le savons.

que des médecins souhaitent s'orienter vers ce type de prescriptions, pourquoi pas, mais, selon moi, cela relève d'une spécialisation

: La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à intégrer dans la formation initiale et continue des médecins des modules relatifs aux droits des femmes, aux stéréotypes de sexe et au respect du corps d'autrui. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la prise en charge de la patientèle et dans la grande cause du quinquennat.

C'est par la formation que nous transformerons les mentalités. Les professionnels de santé ne doivent pas manquer à l'appel. Pour cela, les médecins doivent recevoir une formation sur le repérage des violences sexuelles et sexistes, afin de lutter contre la culture sexiste qui prévaut encore dans de trop nombreux hôpitaux et de soigner correctement les victimes de telles violences.

mais ils peuvent signaler et s'entourer de personnes qui savent.

chargés notamment de la prise en charge des violences faites aux femmes. Ils devront mettre en place un réseau dans les établissements de santé de leur région, avec obligation de formation des médecins qui prennent en charge ces patients, notamment dans les services d'urgence. Tout cela est déjà organisé. Nous avons financé ces dix centres de psychotrauma : j'ai même inauguré celui de Lille voilà quelques mois. Il s'agit de réseaux

notamment la gestion des conséquences sur la santé des pratiques et des modes de vie, attendent les professionnels de santé. Il est donc nécessaire d'adapter la formation des futurs médecins, en leur délivrant un enseignement relatif à la santé environnementale et portant, notamment, sur les effets des polluants locaux ou globaux sur notre santé ; c'est un enjeu majeur de santé publique.

l'occurrence répétée d'une même pathologie. Cela manque cruellement à l'heure actuelle ; il nous faut nous adapter au monde d'aujourd'hui. Les personnels du corps médical sont des interlocuteurs privilégiés pour les citoyens. Ils doivent pouvoir répondre aux inquiétudes. Ils sont écoutés et seront des leviers puissants de progrès. Ils peuvent mettre en garde leurs patients, les appeler à la vigilance. Ils ont un rôle majeur à jouer. Il est nécessaire qu'ils soient formés, afin de pouvoir mieux informer les populations et participer au changement des pratiques dangereuses pour la santé et l'environnement. Les professionnels de santé doivent connaître les risques des expositions aux polluants et les solutions à mettre en place. Un enseignement sur la santé environnementale doit être

Mme Cathy Apourceau-Poly. Madame la ministre, vous êtes sensible aux liens et conflits d'intérêts qui peuvent exister dans le domaine de la recherche, mais vous avez rejeté, à l'Assemblée nationale, un amendement proche de celui-ci, au motif que son adoption conduirait à interdire les stages dans les maisons de santé ou les établissements privés. Nous sommes d'accord sur le fond, et nous espérons donc que vous soutiendrez notre amendement, qui est rédigé différemment. Il y a aujourd'hui une problématique très importante de neutralité économique et commerciale à l'université. Les politiques successives de restrictions budgétaires et le développement des fondations privées en matière d'enseignement supérieur et de recherche ont conduit les universités à se tourner vers les entreprises privées pour financer leurs projets.

sont des médecins sans intérêt » prévaut trop souvent. C'est ainsi que les universités de Strasbourg, d'Amiens ou de Paris VII ont signé entre 150 et 534 conventions avec des laboratoires privés leur fournissant moyens humains et matériels, pour un montant pouvant atteindre 80 000 euros.

Dans le cadre de l'enseignement, ils conditionnent donc leurs étudiants à l'emploi de produits et de marques définis plutôt qu'à celui des substances médicamenteuses contenues dans lesdits médicaments. Cette situation pose forcément plusieurs problèmes majeurs. Elle influence la future pratique des étudiants et elle renforce la porosité entre l'enseignement supérieur et le secteur privé, avec des risques de dérapage : absence d'esprit critique quant à la qualité des produits, influence sur les contenus enseignés,

de la recherche, ne serait-ce que pour appuyer les efforts faits par certains enseignants et étudiants en médecine, qui dénoncent ces pratiques douteuses. Quel

en respectant le principe de neutralité dans toutes ses dimensions, dont la neutralité commerciale, à laquelle vous faites référence. L'indépendance des formations initiale et continue des professionnels de santé est un objectif que nous partageons. Tout ce qui participe à la qualité et à la pertinence des soins, objectifs centraux de l'ensemble des transformations que porte le Gouvernement, est bien sûr au coeur de nos préoccupations. C'est une exigence que nous devons à nos concitoyens. Cependant, il s'agit ici de ce que l'on appelle des formations « professionnalisantes », inscrites dans des environnements d'exercice.

l'alinéa 33, nous proposons que soit également évaluée la qualité des stages proposés aux étudiants dans le cadre de la future réforme du deuxième cycle, au même titre que l'acquisition des connaissances et des compétences ou la construction du projet professionnel, par

De ce point de vue, proposer une évaluation des stages me paraît peu pertinent, d'autant que l'article 2 prévoit déjà l'évaluation du déploiement d'une offre de stages tout au long des études de médecine. Avis défavorable.

Néanmoins, nous proposons d'être encore plus précis en ciblant plus particulièrement les zones sous-denses, d'une part, et les centres de santé en tant que mode d'exercice,

sont une préoccupation majeure pour les parlementaires que nous sommes, sur quelques travées que nous siégions, ainsi que pour les populations concernées. Par conséquent, les étudiants doivent y être particulièrement sensibilisés. De même, faire référence expressément aux centres de santé nous semble intéressant, dans la mesure où ces structures de proximité, encore insuffisamment développées sur le territoire, répondent aux attentes des jeunes professionnels, en permettant notamment le salariat et l'exercice collectif. Quel

La formation initiale des étudiants en médecine, même si les cursus incluent aujourd'hui une formation en gériatrie et en gérontologie, ne met pas suffisamment en avant les atouts objectifs des carrières dans ce secteur. dans ce secteur. Aussi faudrait-il encourager les étudiants, et particulièrement les internes, à réaliser des stages dans des lieux d'accueil de personnes âgées, notamment en Ehpad, afin de les sensibiliser à la question de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes.

au sein de structures diversifiées- maisons de santé, centres de santé, établissements hospitaliers, Ehpad -, sans que la loi ait eu besoin de le préciser. En outre, la notion de « participation à l'activité hospitalière » recouvre nécessairement

dans nos territoires. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a mis l'accent sur le caractère systémique de ces maltraitances institutionnelles. Il est donc important d'inscrire que l'objectif même des études de médecine est de former des soignants à une prise en charge humaine et respectueuse des droits des patients. Cela va mieux en l'écrivant

au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Pour des questions de lisibilité et de cohérence des principes, il ne me paraît pas opportun de l'inscrire sous une formulation différente dans le code de l'éducation.

que le respect de la dignité et du droit des patients fait partie intégrante des études de médecine. Le problème n'est pas tant de l'enseigner que de le mettre en oeuvre.

À côté du savoir scientifique et théorique, il existe un savoir expérientiel, celui des usagers. Le concept de décision médicale partagée, qui a fait l'objet d'une recommandation de l'ARS en 2013, renvoie au processus au cours duquel les médecins et le patient partagent une information médicale pour mieux comprendre les différentes options de soin. Bien entendu, il n'est pas évident ni naturel

mention dans la loi, laquelle n'a pas vocation à définir précisément le contenu des formations en santé. Il semble en outre que l'absence de cette mention n'ait pas empêché les

« Ma santé 2022 ». Cela témoigne de notre volonté de mettre en place des méthodes d'apprentissage complémentaires, afin de permettre aux professionnels de santé de mieux appréhender le patient dans la relation soignant-soigné. La participation des patients à la formation des professionnels, qui est aujourd'hui une pratique peu répandue, même si elle est en train de se déployer dans un certain nombre d'universités françaises, nous paraît importante. Elle est déjà largement pratiquée dans d'autres pays- en Angleterre, au Canada, en Australie, en Italie -, et elle permet de valoriser la connaissance acquise au travers de l'expérience du patient. Il n'y a rien de tel, par

prodigué par les professeurs. L'inscrire dans la loi constitue une base forte pour que les facultés de médecine intègrent ces méthodes à leurs formations et à leurs pratiques d'évaluation. Nous souhaitons également

en matière de santé publique me paraît nettement exagéré. J'en veux pour preuve un article paru récemment, sous la signature du professeur Gentilini, membre de l'Académie de médecine,

En matière de thérapeutique, il est tout de même nécessaire de faire la part des choses et de ne pas confondre traitement et imposture.

en introduisant des orientations liées à la santé environnementale. Eu égard aux nouveaux défis liés à la pollution de l'air, aux perturbateurs endocriniens, à l'absorption de pesticides, aux radiations, à la contamination des milieux, nous devons améliorer la formation des praticiens

l'importance des plans nationaux santé-environnement, mais il s'agit d'accompagner et de renforcer ce mouvement, et de répondre aux nombreuses inquiétudes, justifiées, de nos concitoyens face à la multiplication des pathologies dites environnementales. Inscrire la dimension de la santé environnementale dans les orientations pluriannuelles prioritaires et dans la formation continue des professionnels de santé me paraîtrait constituer

Avec l'article 2 , il s'agit de modifier l'article du code de l'éducation qui fixe les principes et les objectifs généraux des études de médecine.

d'une confusion dans les objectifs des études de médecine ; celles-ci doivent avant tout servir à former de futurs médecins et non à répondre aux carences territoriales de l'offre de soins. Je crains que nous n'ayons pas encore toutes les garanties quant au déploiement d'une offre de stages de qualité dans les zones sous-denses, du fait, notamment, du manque de maîtres de stage. En attendant que cette condition soit remplie, la commission ne juge pas opportun de dégrader potentiellement l'encadrement de certains étudiants, et donc la qualité de leur formation.

pour accueillir, au cours d'une même année, l'ensemble d'une promotion- à peu près 9 000 étudiants, toutes spécialités confondues

Il est quelque peu paradoxal que le problème de la médecine de ville soit la médecine de campagne Il est nécessaire d'attirer des médecins dans nos campagnes, où les Français expriment largement, dans de nombreux scrutins et sur de nombreux ronds-points,

Nous avons la faiblesse de penser que la mesure que nous avons proposée est d'un autre niveau. Elle prolonge le sillon incitatif, mais en le creusant de façon plus volontariste et plus rapide.

le nombre de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles. Les territoires parvenant à recruter des jeunes médecins sont ceux qui se montrent particulièrement actifs en termes de création de maisons de santé pluriprofessionnelles- je pense notamment à l'Aveyron, exemplaire sur ce plan.

Cet amendement vise à permettre à un étudiant en médecine de troisième cycle de réaliser son stage obligatoire d'internat dans son département d'origine, même s'il poursuit ses études dans une autre région. En effet,

études, d'un autre département, d'une autre région, d'une autre agence régionale de santé, et ont aujourd'hui l'obligation de faire leur stage dans le périmètre de leur université, soit le Grand Est. Sans accord pédagogique et sans possibilité de transaction financière entre les agences régionales de santé- le maître de stage étant rémunéré -, les Axonais qui étudient à la faculté de médecine de Reims ne peuvent pas faire leur stage d'internat dans l'Aisne. Quel

existe depuis de nombreuses années. De tels stages sont même parfois nécessaires à la réalisation de certains parcours de formation. Très appréciés des étudiants, ils font l'objet de modalités de financement spécifiques, dans le cadre du financement du troisième cycle, afin que la contrainte budgétaire constitue un frein minimal à leur mise en oeuvre. Je reconnais néanmoins que l'on doit pouvoir encore simplifier et améliorer les choses. La réforme du troisième cycle a d'ailleurs conforté ces stages en ouvrant la possibilité aux étudiants de demander deux stages dans une région différente

décidément faire faire beaucoup de choses aux étudiants en médecine : au cours du deuxième cycle, ils devraient participer à des échanges internationaux, faire des stages de médecine générale, effectuer des stages

L'article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet que, dans le cadre du parcours de soins d'un patient atteint d'une affection de longue durée, le médecin traitant puisse prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. de prescription d'activité physique adaptée par le médecin traitant a été déclinée par le décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée. Cette pratique du « sport sur ordonnance » concerne 10 millions de personnes souffrant d'ALD telles que la maladie de Parkinson, certains cancers, le diabète, etc. Elle permet d'améliorer leur condition physique, de diminuer la dépendance du système de soin à l'allopathie, de réduire les risques de récidive et de réhospitalisation.

de cet amendement souhaitent inciter les médecins des réseaux de santé, des centres de santé ou encore des maisons de santé à se former pour pouvoir accompagner un étudiant en médecine lors d'un stage.

même si ce n'est pas obligatoire. Il n'est donc pas nécessaire de le prévoir expressément dans la loi. J'émettrai en outre deux réserves sur cet amendement. La première réserve porte sur le ciblage des structures. Il pourrait également être intéressant,

Cela ne signifie pas qu'il faudrait prévoir des objectifs d'accueil de stagiaires également pour ces structures ; simplement, il n'est pas nécessairement opportun de viser certaines structures plutôt que d'autres, car cela peut brouiller le message envoyé aux étudiants et aux acteurs de santé. La seconde

Cela nécessite, en particulier, de prévoir ces stages dans les maquettes de formation, mais également de former suffisamment de maîtres de stage. À ces conditions, les étudiants pourront faire des stages dans tout type de structure ambulatoire dans des conditions d'encadrement satisfaisantes, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant.

L'augmentation du nombre d'étudiantes et d'étudiants en médecine et de futurs infirmiers pose évidemment la question du nombre de maîtres de stage en mesure de les accueillir. Concernant la médecine générale, voilà quelques semaines, le Syndicat national des enseignants de médecine générale a publié des chiffres annuels très encourageants en matière de maîtrise de stage. Le nombre de maîtres de stage des universités progresse pour la troisième année consécutive au sein de la filière universitaire de médecine générale, pour dépasser le cap symbolique des 10 000.

Pourtant, les textes prévoient le suivi obligatoire d'un stage d'initiation à la médecine générale en cabinet libéral, en maison de santé ou en centre de santé pendant l'externat. Ce stage n'est pas effectué partout, en raison d'un déficit de maîtres de stage, mais aussi d'un manque de volontarisme des unités de formation et de recherche en santé. Il n'en constitue pas moins une étape essentielle pour découvrir une spécialité méconnue et trop souvent dévalorisée au sein d'un second cycle qui demeure fortement hospitalo-universitaire. Cet amendement vise à faciliter l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycles de médecine, afin de diversifier et de multiplier les lieux de stage, ce qui permettra e l'orientation de davantage d'étudiants vers la médecine générale et les territoires sous-dotés.

En premier lieu, il tend à compléter la base législative du code de la santé publique ouvrant la possibilité aux étudiants en médecine de réaliser des stages extrahospitaliers, pour étendre celle-ci aux étudiants de deuxième cycle sans l'inscrire dans le code de l'éducation. Cela signifie qu'il sera possible aux étudiants d'effectuer de tels stages sur la base du volontariat, même si le code de l'éducation ne le prévoit pas expressément. auteurs de cet amendement soulèvent une question pertinente quant aux modalités concrètes de réalisation de ces stages, en prévoyant un encadrement au niveau législatif de l'agrément des maîtres de stage. À l'heure actuelle, ce régime n'est défini qu'au niveau réglementaire, ce qui est sans doute insuffisant. Il est donc proposé de déterminer cet encadrement à droit constant, tout en fixant le principe d'une formation obligatoire. L'avis de la commission

L'enjeu premier réside tout autant dans le processus de formation des praticiens à la maîtrise de stage que dans l'émergence de candidatures à l'agrément de lieux de stage répondant aux critères pédagogiques requis pour accueillir et former les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine. Ces deux processus sont complémentaires, c'est dans ces deux directions que toutes les mesures susceptibles de faciliter la maîtrise de stage doivent être envisagées, avec le souci permanent de préserver la qualité de l'encadrement et de la formation. Ces mesures relèvent actuellement du niveau réglementaire et doivent être en permanence étroitement concertées. C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à ce que des options soient ainsi préemptées au niveau de la loi, ce qui rendrait leur éventuelle adaptation beaucoup plus compliquée. Nous sommes néanmoins bien

des territoires. Leur statut est particulier, puisqu'ils sont toujours des étudiants, mais des étudiants dont la formation est déjà bien avancée et qui peuvent réaliser toute une série d'actes médicaux. Malheureusement, la formation des internes en médecine est trop tournée vers le secteur hospitalier. Si les stages en cabinet médical ont été rendus possibles récemment, ils sont encore trop peu fréquents et il est nécessaire d'augmenter le nombre de maîtres de stage. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à imposer aux étudiants en médecine de troisième cycle

Dans le cadre de la refonte des études médicales, les étudiants de troisième cycle sont appelés à réaliser des stages dans divers services hospitaliers ou en ambulatoire. Aujourd'hui, tous les étudiants de troisième cycle n'ont pas la possibilité de faire leurs stages au sein d'associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, ce qui est regrettable. Le présent amendement prévoit que les médecins généralistes exerçant dans des associations de soins non programmés et de permanence de soins ambulatoires, tels que les 1 300 médecins

par tout médecin généraliste aux internes qui réaliseraient leur stage sous son encadrement. L'accueil d'étudiants au sein des associations est donc tout à fait possible en l'état actuel du droit. Cet amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

Cet amendement vise à autoriser, à Mayotte, les étudiants de troisième cycle de médecine générale à effectuer une partie de leurs stages pratiques dans des dispensaires. Mayotte

du code de la santé, lequel impose actuellement aux étudiants de troisième cycle d'effectuer leurs stages auprès de médecins généralistes agréés. Au regard de l'urgence sanitaire dans certains territoires, du manque criant de spécialistes et des délais d'attente,

du projet de loi, dont la portée semble par ailleurs plus large, dans la mesure où il autorise les étudiants de toutes spécialités à effectuer leurs stages auprès de praticiens libéraux, sans restriction territoriale.

professionnalisant de trois mois, le clinicat. Les critères d'évaluation de ce stage intègrent, notamment, la capacité de l'étudiant à concevoir et à mettre en oeuvre un projet de soin de manière autonome, sous supervision du maître de stage. L'autonomisation de l'étudiant dans la gestion d'une prise en charge induit une augmentation de la patientèle, ce qui n'a jamais posé de problème pour les étudiants en médecine stagiaires. Or le cadre juridique actuel n'autorise pas l'augmentation de l'activité

L'interdiction de l'accroissement de l'activité rémunérée à l'occasion d'un stage a une finalité protectrice des patients comme des étudiants. Le code de la santé publique dispose que les actes remboursés par l'assurance maladie sont réputés être accomplis par des professionnels diplômés.

Si, une fois encore, nous ne sommes pas opposés par principe aux ordonnances, il est regrettable que le texte de loi ne retranscrive que trop sommairement les recommandations du rapport du professeur Uzan, dont il semble pourtant s'inspirer largement. Dès lors, cet article 3 baigne dans un flou artistique, qu'il s'agisse du fond de la réforme envisagée ou des moyens qui lui seront dédiés. Nous le regrettons.

Si le DPC doit être l'une des composantes de la recertification, comme l'a indiqué la direction générale de l'offre de soins devant la commission des affaires sociales, il apparaît clairement que des moyens supplémentaires devront être prévus. Qu'en est-il, madame la ministre ? Enfin, je me permets d'attirer votre attention sur un autre point : la procédure de recertification devra être bien plus simple que le DPC actuel. Aujourd'hui, rien n'est fait pour faciliter une démarche aussi essentielle qu'exigeante. La parole

la recertification. Beaucoup souhaitent que le DPC soit un mode de recertification ou intervienne dans les possibilités de recertification.

L'objectif est de maintenir un haut niveau de compétences tout au long de la carrière professionnelle. Or la formation continue obligatoire des médecins est essentiellement assurée par l'industrie pharmaceutique, qui peut ainsi les inciter à prescrire ses propres produits.

à but lucratif sans lien avec l'industrie, tels que les structures émanant de centres de lutte contre le cancer, pour reprendre l'un des exemples que vous aviez cités. Le sous-amendement

consulter. En l'absence d'égalité de traitement des médecins devant la recertification de leurs compétences, s'établirait un système comportant deux catégories de professionnels : ceux dont les connaissances seraient systématiquement contrôlées et certifiées et ceux qui auraient le choix de se soumettre ou non à cette mesure.

que j'ai compris, les acteurs qui mettront en oeuvre la certification pourraient être notamment la Haute Autorité de santé, les ordres et les conseils nationaux professionnels,

au détriment d'autres et de leur attribuer un rôle précis, alors que les arbitrages ne sont pas rendus. C'est précisément pour permettre à la concertation d'approfondir ces questions que nous avons choisi de procéder par ordonnance. La démarche de préparation des arbitrages et de rédaction de l'ordonnance et des textes réglementaires

est à Mme la ministre. La loi prévoit que les professionnels de santé du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique sur le handicap.

Ces violences ont des conséquences graves sur la santé des femmes, et la libération de leur parole permettrait sans doute de diagnostiquer et de traiter des pathologies dont elles peuvent souffrir. Or la détection des violences sexuelles par les professionnels de santé fait défaut, en raison notamment du manque de formation du corps médical à ces questions. Il est urgent, à mon sens, de remédier à cette lacune. Par ailleurs, des études récentes ont mis en lumière de nombreux cas de violences gynécologiques et obstétricales, d'infantilisation ou de défiance à l'égard de la souffrance des femmes de la part de professionnels de santé. Ces situations ne doivent plus durer. Les femmes doivent pouvoir franchir sereinement le seuil des hôpitaux et des cabinets médicaux. En outre, en matière de droits sexuels et reproductifs, certains professionnels peuvent se montrer insuffisamment formés à la pratique des actes et à l'accueil des femmes pour des cas d'IVG ou de suivi des contraceptifs, ce qui peut mener à des situations compliquées et douloureuses pour les femmes. C'est pourquoi nous proposons que la formation continue

est plus efficace que les traitements conventionnels, avec moins d'effets secondaires ; dans d'autres, les plantes peuvent être utilisées en association avec les médecines conventionnelles. En particulier, le recours aux plantes est une réelle opportunité pour réduire la consommation d'antibiotiques, particulièrement élevée en France, ce qui pose problème à l'heure où les antibiorésistances sont une menace majeure.

L'enjeu est particulièrement important dans les outre-mer, où l'usage des plantes et le recours aux médecines traditionnelles sont très répandus. Afin de garantir un meilleur accès à l'information des patients et une réponse à leur demande de soins à base de plantes, les auteurs de l'amendement proposent de prévoir dans la loi la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social à la santé par les plantes. Eu égard à la faible intégration des plantes dans notre système de soins, inscrire cette formation dans la loi paraît essentiel pour envoyer un signal fort ! Quel

La faible place des plantes dans notre système de santé est, je le répète, très regrettable, parce que nous nous privons de thérapies efficaces, mais aussi parce que les professionnels de santé ne peuvent pas, dans bien des cas, prendre en compte les potentielles interactions médicamenteuses. Dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, les professionnels qui souhaitent mettre en place des protocoles utilisant les plantes rencontrent des difficultés, alors même que certains produits végétaux sont plus efficaces que les thérapies

mais qui est insuffisamment connu, comme l'ont indiqué les organisations étudiantes que nous avons rencontrées. Ainsi, en dix ans, seuls 2 800 contrats ont été signés par des étudiants et des internes en médecine, avec une montée en charge progressive, puisque ce sont plus de 550 contrats qui ont été conclus en 2017-2018. Pourtant, cet outil incitatif à l'installation de jeunes praticiens en zones sous-dotées aurait dû constituer une réponse plus efficace au problème des déserts médicaux. Madame la ministre, avez-vous des éléments d'évaluation et de compréhension qui pourraient expliquer les raisons du peu d'attractivité de ce dispositif ?

de l'absence d'emploi pour le compagnon ou la compagne. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur les conséquences concrètes des lois que nous votons ici, ou, pour le coup, que le groupe CRCE ne vote pas. Comment ignorer que la réduction des dépenses publiques a un impact dans nos territoires ? D'où la situation que nous connaissons aujourd'hui : de jeunes médecins hésitent, assez légitimement, à s'installer dans des endroits où il ne reste plus grand-chose. Et dire que le Gouvernement prévoit encore la suppression de 120 000 fonctionnaires ... C'est très alarmant et cela devrait nous faire faire réfléchir. Rendre le contrat d'engagement de service public plus contraignant, en supprimant la possibilité pour les signataires de modifier leur lieu d'exercice ou en introduisant un classement des candidatures, nous paraît contre-productif. En revanche, nous approuvons le fait que le CESP soit élargi aux Enfin, madame la ministre, pourquoi ne pas réfléchir à des aides pour trouver un logement, des aides pour les transports, etc., autant de petits plus suggérés par les jeunes médecins que nous avons rencontrés en vue d'améliorer réellement ce dispositif ? La parole

à diplôme hors Union européenne. Tout ce qui va dans le sens d'une meilleure répartition des praticiens sur le territoire mérite d'être soutenu. Néanmoins, cela apparaît nettement insuffisant au regard des besoins, ce qui traduit la légèreté avec laquelle ce projet de loi traite l'enjeu des déserts médicaux. Le principe du CESP est simple : il s'agit d'un contrat par lequel les étudiants en médecine s'engagent à s'établir dans une zone dans laquelle la continuité des soins est menacée ou à choisir une spécialité moins représentée, en contrepartie d'une allocation mensuelle de 1 200 euros versée durant leurs études. Ils devront s'installer pendant un nombre d'années égal à celui durant lequel ils auront perçu l'allocation, et pour deux ans minimum. Aussi attractif qu'il puisse paraître, ce dispositif ne suffit pas. Seuls 8 % des étudiants de seconde année ont signé un contrat pour 2016-2017, soit 486 étudiants. Nous touchons là du doigt les limites, pour ne pas dire plus, des dispositifs incitatifs. Il est urgent de mettre en place des mesures claires, plus volontaristes, de régulation à l'installation des médecins ; je pense, par exemple, au conventionnement sélectif en fonction du niveau de dotation des territoires en professionnels de santé.

Voilà un dispositif intéressant, qui poursuit sa montée en charge et commence à produire ses effets. Son principe est simple : en contrepartie d'une allocation mensuelle, les étudiants s'engagent à s'installer à l'issue de leur formation en zone sous-dense. Depuis sa mise en place en 2010, à la suite de l'adoption de la loi HPST, ce sont plus de 2 800 contrats d'engagement de service public qui ont été signés, dont 550 pour l'année 2017-2018, traduisant une nette progression. Si un tel dispositif doit bien évidemment être développé- l'extension aux praticiens à diplôme hors Union européenne qui est prévue dans ce projet de loi est une bonne mesure -, il est nécessaire d'en améliorer encore le fonctionnement.

À cet égard, le délai de deux ans prévu par la loi pour conserver sur la liste des lieux d'exercice proposés à la signature du CESP ne paraît pas suffisant pour permettre aux étudiants d'envisager sereinement leur projet professionnel. Au-delà des nécessaires perfectionnements du dispositif, je veux le souligner encore une fois, c'est tout le panel des outils destinés à mettre fin aux déserts médicaux qu'il convient d'étendre. Nous en avons parlé, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une politique plus volontariste en la matière : il faut redonner à ces territoires l'attractivité qu'ils méritent. La parole

des jeunes médecins et dentistes dans les déserts médicaux, en contrepartie d'une allocation mensuelle versée lors de leurs études. Notre groupe y est bien sûr

nous le constatons, ils ne sont pas suffisants, puisque, au fil des années, les inégalités territoriales s'accroissent, avec des densités médicales extrêmement différentes : de 1 à 3 pour les généralistes, de 1 à 8 pour les spécialistes,

au cours de la séance, examiner des amendements allant en ce sens. C'est tout à l'honneur du Sénat que de se pencher sur le volet territorial de ce texte, plus que ne l'a fait, notamment, l'Assemblée nationale. Nous avons déjà amélioré le texte hier soir en adoptant un amendement visant à rendre obligatoires les stages en troisième cycle.

C'est l'un des leviers pour faire en sorte que, partout sur le territoire, des médecins se déploient, justement parce qu'ils sont issus de territoires situés en zone sous-dense et de milieux défavorisés.

que davantage d'étudiants issus des milieux ouvriers ou de l'agriculture puissent devenir médecins à leur tour, comme autrefois, car ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est

85 % d'entre eux seulement ont été signés, soit 550 contrats. Dans ce contexte, ajouter une condition pour le bénéfice du CESP pourrait entraver le déploiement de cet outil, que nous devrions au contraire encourager. Nous pourrons, je pense, et je l'espère, en reparler si, un jour, il y avait plus de demandes que de contrats offerts. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable

payer des études dans une ville universitaire pendant deux ans, avec un risque d'échec majeur. Cette diversification des profils dans l'entrée des études de médecine vise aussi

La liste actuelle des lieux concernés proposée par le Centre national de gestion, sur suggestion des agences régionales de santé, les ARS, concerne, pour sa très grande majorité, des centres hospitaliers. Or, même dans des zones qui ne sont pas considérées comme des zones sous-dotées, les établissements sociaux et médico-sociaux peinent à recruter des médecins. La nécessité par ailleurs de décloisonner secteur médico-social et sanitaire au profit d'une population vulnérable est indispensable. L'objet de cet amendement est d'ouvrir le bénéfice de l'exercice médical des praticiens signataires d'un contrat d'engagement de service public aux établissements sociaux et médico-sociaux, quel que soit leur lieu d'implantation et non aux seuls établissements situés en zone sous-dotée.

fait référence à la localisation géographique des lieux d'exercice, et non aux structures de soins auxquelles ils seraient rattachés. En second lieu, rien dans la rédaction de l'article L. 632-6 du code de l'éducation n'empêcherait que ces lieux d'exercice soient situés en établissement médico-social. Il n'est donc pas utile de le préciser dans la loi, à moins de mentionner également qu'ils peuvent être situés en établissements de santé, mais nous rencontrerions alors le problème inhérent à toute énumération législative : le risque d'oubli, avec les conséquences contre-productives qui pourraient en découler.

préciser les raisons pour lesquelles les lieux d'exercice sont principalement situés dans des centres hospitaliers. Faute d'un retrait, la commission serait obligée d'émettre un avis défavorable

à des médecins de s'installer dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante, quel que soit le mode d'exercice, qu'il soit libéral, hospitalier ou intervenant dans le secteur médico-social,

Les associations étudiantes que j'ai rencontrées m'ont toutefois fait part des insuffisances de ce dispositif. Il est en effet possible qu'un étudiant ayant signé un CESP au cours de sa formation ne bénéficie plus de la même liste de lieux d'exercice à l'issue de son cursus si le zonage évolue entre-temps.

Or le CESP constitue un levier efficace, qu'il convient de mobiliser davantage au profit des territoires en difficulté. Pour preuve, 90 % des signataires se sont installés en activité libérale, et une grande majorité des CESP signés concernent des médecins généralistes. Cet amendement vise à répondre à une demande pragmatique formulée par les internes de médecine générale avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger ; son adoption permettra aux signataires de se projeter dans un territoire, d'y construire leur projet personnel, sans s'inquiéter de l'évolution du zonage. En pratique, il tend à rendre le dispositif plus efficace en alignant la durée du bénéfice du CESP en cas d'évolution du zonage sur la durée de l'internat de médecine générale, c'est-à-dire trois années. objet de conforter les objectifs poursuivis à l'article 4, car il vise à sécuriser davantage les CESP. Une telle mesure contribuera sans nul doute à la montée en puissance souhaitable de ce contrat. Pour rappel, quelque 3 125 contrats ont été signés depuis 2010, et 500 signataires se sont déjà installés.

aux étudiants et internes en médecine en échange d'un engagement à exercer dans des zones sous-dotées. Après six ans de mise en place, le dispositif des CESP monte en puissance, avec 521 postes ouverts en médecine pour l'année 2018, et apporte par là même une réponse prometteuse pour lutter contre la désertification médicale. Malgré ce bilan positif, le dispositif des CESP se heurte à plusieurs freins empêchant un déploiement plus important, notamment au regard des mises à jour régulières des zonages par l'ARS, qui définit les zones où un signataire d'un CESP est éligible pour l'installation. Ainsi, certaines zones éligibles au moment de la signature ne le sont plus lors de l'installation, ce qui oblige le signataire à repenser en totalité son projet d'installation au dernier moment, voire le conduit, dans certains cas, à une rupture du contrat. Si le projet de loi prévoit que le Centre national de gestion maintienne sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins dans les deux ans précédant la publication de la liste, ce délai ne semble pas suffisant pour se prémunir véritablement des problèmes constatés. Aussi, nous proposons que cette liste des lieux d'exercice soit maintenue pendant trois ans, au lieu des deux ans prévus dans le texte actuel. Le CESP est une mesure incitative, car il favorise l'installation des jeunes médecins dans les zones sous-denses. Il répond aux besoins des territoires et contribue à lutter contre la désertification médicale. Notre amendement a pour objet de le consolider. La

très positifs sur l'installation des médecins dans ces zones en difficulté. Le fait d'inciter, et non pas d'obliger les médecins à s'installer dans ces zones pendant une période

n° 298. Les contrats d'engagement sont un outil pertinent pour conduire des futurs praticiens de santé à se fixer dans des territoires sous-dotés, et ainsi transformer une incitation en projet concret. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 20

Il ressort donc de cette formulation que le CESP peut, dans certains cas, perdre de son intérêt ou, à tout le moins, léser les étudiants en médecine ou en odontologie. Pour cette raison, nous vous demandons de prolonger d'un an la garantie du maintien des zones sous-denses dans le dispositif, afin d'assurer l'effectivité du contrat d'engagement jusqu'à trois ans. Ainsi, un interne de médecine générale commençant son internat sera certain de la zone dans laquelle il pourra s'installer à la fin de son cursus. La parole

L'article 4 comporte une disposition visant à sécuriser le choix du futur lieu d'exercice des bénéficiaires d'un CESP. En effet, les zones sous-denses ne sont pas figées il se peut qu'un étudiant élabore son projet professionnel dans un territoire qui n'est plus, au terme de ses études, considéré comme une zone sous-dotée. Le projet de loi prévoit la possibilité de maintenir sur la liste des lieux prévoit la possibilité de maintenir sur la liste des lieux d'exercice qui sont proposés aux signataires à l'issue de leurs études des lieux qui y figuraient deux ans auparavant, mais qui ne sont plus considérés comme des zones sous-denses. Cette mesure a pour objet de sécuriser les projets professionnels des étudiants. Ces amendements de la fonction publique hospitalière, le CNG, a la possibilité de conserver sur la liste des lieux d'exercice proposés ceux qui y figuraient trois ans auparavant, et non plus deux. Il s'agirait ainsi de s'aligner sur la durée de l'internat. Je comprends la philosophie de ces amendements. Pour autant, la commission émet deux réserves. Tout d'abord, l'article 4 prévoit que le choix du futur lieu d'exercice ne se fait plus nécessairement au cours de la dernière année des études il pourrait se faire au début du troisième cycle, auquel cas les amendements proposés auraient moins de sens. Ensuite, et surtout, la durée de l'internat n'est pas nécessairement de trois ans pour toutes les spécialités.

La directive de 2005, modifiée en 2013, ne prévoit pas de changement de durée pour le diplôme d'études spécialisées- le DES -de médecine générale, qui est et reste fixée à trois ans.

Ce décret n'est en effet applicable qu'aux spécialités comprenant une phase de consolidation et supposant, donc, au moins quatre ans de formation. Or j'observe que la question du passage de trois à quatre ans du DES de médecine générale constitue depuis quelques années un serpent de mer du débat public.

de la maquette à quatre ans ne pourrait être envisagé que dès lors que les objectifs visés par une telle mesure et les conditions de sa mise en oeuvre dans le cadre du nouvel équilibre de la maquette en huit semestres feraient l'objet d'un consensus de tous les acteurs. faudrait que les conditions de sa soutenabilité, notamment sur le plan pédagogique, au regard du nombre de maîtres de stage disponibles, soient réunies. Cela implique, pour le Gouvernement, que la concertation

il y a besoin de répondre à l'attente des médecins, des élus et, surtout, de nos concitoyens. Je pense que la solution proposée au travers de ces amendements est une réponse pragmatique, qui, encore une fois, n'est pas coercitive- il faut prononcer le mot -pour les étudiants. On leur tend la main et on vous tend la main, madame la ministre. Il faut que nous travaillions ensemble. Encore une fois, ces étudiants ne seront pas

une simplification et rendre ces aides plus attractives et plus lisibles pour les jeunes médecins. Ce travail est en cours et devrait m'être remis en juillet Madame Imbert, vous affirmez que la professionnalisation fait partie intégrante de la formation. C'est

42, selon lequel « pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région ».

relatif aux libertés d'exercice et d'installation des médecins, afin de faire apparaître la nécessité, pour les médecins, de prendre en compte le principe d'égal accès aux soins.

a véritablement pris la mesure du problème de l'accès aux soins et qu'il entend marquer son attachement aux principes constitutionnels qui fondent notre pacte social. La parole

entre les médecins et l'assurance maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. En l'absence d'accord, il est proposé de mettre en place un système de conventionnement sélectif, pour limiter les installations de médecins dans les zones surdotées. Un dispositif similaire est depuis longtemps appliqué à d'autres professions, chaque fois avec des résultats satisfaisants. J'ajouterai que la Cour des comptes préconise d'étendre, dans les zones en surdensité, surdensité, le conventionnement conditionnel à toutes les professions, y compris aux médecins, pour mieux équilibrer la répartition des professionnels sur le territoire. Selon la Cour, la régulation des installations est une nécessité pour obtenir un rééquilibrage des effectifs libéraux, en fonction des besoins de santé des populations sur le territoire, et elle peut être recherchée sans remettre en cause la liberté d'installation, en instituant un conventionnement individuel généralisé à l'ensemble du territoire. Si l'on veut lutter efficacement contre la désertification médicale, il est essentiel de mobiliser l'ensemble des leviers, notamment ceux qui ont fait leurs preuves. Tel est l'objet de cet amendement.

des médecins libéraux, afin d'assurer une meilleure répartition sur le territoire et de lutter contre la désertification médicale. proposons de conditionner le conventionnement d'un médecin à la cessation d'activité d'un autre médecin exerçant dans la même zone. Je rappelle tout de même que la Nation prend en charge la formation des médecins, un coût qui avoisinerait 11 540 euros par étudiant chaque année. Je rappelle aussi que l'État assure, bien sûr, les revenus des médecins à travers l'assurance maladie. Or la situation est extrêmement grave.

Plus alarmant encore, les difficultés d'accès aux spécialistes que sont les gynécologues, les ophtalmologistes et les pédiatres concernent jusqu'à 21 millions de nos concitoyens. La question est simple

En lien avec la position adoptée en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, cet amendement tend à poser le principe d'un renvoi aux négociations conventionnelles entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie, leur laissant le choix des moyens, que ce soit un conventionnement sélectif, individuel ou autre, pour aboutir à une solution négociée de nature à traiter efficacement les déserts médicaux. En outre, il vise à mettre en place un système dit de conventionnement individuel sur l'ensemble du territoire, applicable uniquement aux médecins entrant en exercice : les agences régionales de santé, ou ARS, fixeraient le nombre cible de postes de médecins conventionnés, généralistes et spécialistes, dans chaque région et chaque département, en fonction de critères de densité. Dans chaque région et département, les médecins commençant à exercer ne pourraient accéder au conventionnement à l'assurance maladie que sous réserve d'entrer dans les effectifs ciblés. Cette mesure peut sembler moins efficace qu'un conventionnement individuel

En tant qu'élu, les sollicitations sont quotidiennes ; en tant que sénateur, notre devoir est de représenter les territoires. Or les citoyens crient chaque jour leur détresse face à cette inégale répartition de l'offre de soins. C'est l'égalité des territoires qui est en jeu, ainsi que notre pacte républicain Madame la ministre, vous affirmez qu'avec la suppression du la France formera 20 % de médecins supplémentaires. Mais quelle garantie avons-nous qu'ils s'installeront dans les zones déficitaires et dans nos villages ?

le contenu de la proposition de loi, défendue par notre collègue Guillaume Garot à l'Assemblée nationale, visant à instaurer un conventionnement sélectif, pour lutter efficacement contre la désertification médicale. Avec cet amendement, notre objectif est de limiter l'aggravation de ce phénomène, en étendant aux médecins libéraux, à titre expérimental, un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà, cela a été dit par plusieurs de mes collègues, pour plusieurs autres professionnels de santé. L'adoption d'un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement des dispositifs d'incitation à l'installation dans les zones sous-dotées, mis en place dans le cadre du projet de loi de financement

négociation conventionnelle entre l'assurance maladie et les médecins, pour définir les conditions dans lesquelles ces derniers participent à la réduction des inégalités d'accès aux soins et, le cas échéant, les mesures de limitation d'accès au conventionnement dans les zones surdotées.

la négociation des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du [code de la sécurité sociale] doit porter, pour assurer l'offre de soins, sur le conventionnement à l'assurance maladie des médecins libéraux dans les zones définies par les agences régionales de santé, en application en application des 1° et 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ». Ensuite, si les partenaires ne parviennent pas à se mettre d'accord dans un délai d'un an, un dispositif de conventionnement sélectif est prévu, à titre expérimental, pour une durée de trois ans en zones surdotées, selon le principe d'une arrivée pour un départ. Cela permettrait de réorienter progressivement les médecins vers des secteurs intermédiaires et sous-denses. Ce dispositif a prouvé son efficacité pour les infirmiers, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes. Nous connaissons tous les chiffres : les installations en zones surdenses ont largement diminué et celles qui concernent des zones très sous-dotées ont augmenté. Je ne comprends pas pourquoi les médecins ne pourraient pas faire l'objet de dispositions similaires, sous réserve de certaines adaptations, bien entendu, afin de prendre en compte le rôle central qu'ils jouent

n° 423. Cet amendement est le dernier que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a souhaité proposer sur ce projet de régulation des installations des médecins je remercie mes collègues commissaires, en particulier Michel Vaspart, de l'avoir également repris. En 2015, le Sénat avait adopté un dispositif ambitieux, faisant référence à la négociation conventionnelle et à la limitation d'accès au conventionnement comme mesure de régulation de l'offre de soins. Dans une logique de compromis, mes chers collègues, je vous propose de voter le premier membre de ce dispositif, à savoir un renvoi simple aux négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les médecins pour déterminer les conditions dans lesquelles ces derniers participent à la résorption des déserts médicaux. À mon sens, c'est le minimum que puisse faire le Sénat pour adresser un signal politique fort aux élus locaux et aux citoyens, qui nous demandent la mise en place de mesures ambitieuses pour l'accès aux soins. La parole

lors de la seconde, j'ai vu poindre le sujet de la désertification médicale ; lors de la troisième, madame la ministre, les 300 maires

désertification médicale, cet amendement vise à transposer aux médecins libéraux le mécanisme de conventionnement applicable actuellement aux infirmiers libéraux. Cette convention expérimentale, conclue d'ici au 1juillet 2020 et applicable pour une durée de cinq ans, permettrait à la fois de conforter les mécanismes incitatifs pour l'installation dans les zones sous-dotées et d'instaurer un conventionnement sélectif, afin de limiter l'installation dans les zones surdotées. L'impact de la convention est évalué par les parties prenantes dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d'évaluation est publié avant la signature de la convention ; un autre est publié au plus tard le 1 janvier 2023

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris